La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

et garantira l'adhésion des collectivités locales et des Français. Plutôt qu'une répartition décidée par la région, dont le texte entend faire le grand répartiteur des droits à construire, nous avons souhaité que les territoires puissent fixer, en responsabilité, leurs propres objectifs dans le respect d'une orientation générale.

En particulier, ils devront prendre en compte l'existence de projets d'intérêt particulier pour les communes ou les projets d'intérêt commun pour le bassin, les besoins de revitalisation rurale ou d'habitat, ou encore les efforts déjà réalisés

la commission, la notion de sobriété foncière n'est pas définie dans la loi. Elle renverrait évidemment à une exigence de gestion économe de l'espace, mais ne permettrait pas de clarifier ni de modifier le droit existant et, donc, de soutenir l'ambition de lutte contre l'artificialisation des sols, telle que nous l'avons d'ores et déjà définie.

soit décidée à un échelon plus proche des élus compétents en matière d'urbanisme. Le Sraddet n'est pas un document d'urbanisme, et son élaboration est souvent perçue comme une grand-messe, où tous les arbitrages sont déjà rendus avant même que les maires puissent faire valoir leur point de vue.

Je partage évidemment l'objectif qui consiste à revenir au système de territorialisation au niveau régional. Cependant, l'amendement n° 1759 rectifié ne vise que la consommation d'espace naturel, agricole et forestier, et non l'artificialisation des sols.

organise ce dialogue autour de l'application territorialisée et différenciée des objectifs au niveau des SCoT, en garantissant la prise en compte des différents enjeux auxquels sont confrontés les collectivités territoriales. Cette répartition des efforts entre collectivités devra

La parole est à M. Stéphane Demilly. L'article 49 intègre l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionaux. S'il est nécessaire et légitime que la lutte contre l'artificialisation des sols et la réduction de la consommation des espaces naturels soient intégrées dans les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,

le bassin versant de la Seine avec le réseau fluvial du nord de la France et du Benelux. Pour lever toute ambiguïté, cet amendement tend à indiquer que les projets d'envergure régionale ou nationale dont les travaux ont déjà commencé, ce qui est le cas du canal Seine-Nord Europe, seront décomptés de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. La non-prise en compte des grands projets sera évidemment à double sens : l'artificialisation qui en résulte ne sera, certes, pas prise en compte dans le volume des années à venir, mais elle ne le sera pas non plus dans le volume des dix années précédentes. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant

de même un peu en contradiction avec l'ambition que porte le Gouvernement au travers du plan de relance, à savoir la réindustrialisation des territoires et la poursuite, voire l'accélération des investissements dans les entreprises industrielles françaises. amendement a donc pour objet d'aménager les dispositions pour les projets en cours et les projets de réindustrialisation des territoires.

Pour réussir cette territorialisation, nous avons souhaité définir les critères selon lesquels cette répartition entre collectivités s'organisera. Parmi ces critères, nous avons retenu les besoins en logement, le potentiel foncier, les besoins de développement rural, les efforts déjà réalisés ou encore les projets d'intérêt communal ou intercommunal particulier. Je signale à M. Salmon qu'il ne s'agit pas de dérogations personne ne sera dispensé de cibles. En revanche, ces critères permettront de moduler les efforts réalisés par tel ou tel territoire au vu de ses spécificités. C'est ainsi que la commission a traduit l'impératif de différenciation. Je suis donc très défavorable à leur suppression. L'amendement n°

au titre de l'artificialisation. La rédaction que nous avons retenue et les amendements que nous avons adoptés le satisfont déjà, car ces projets ne seront pas pris en compte au niveau des SCoT et des documents locaux. Je suis donc défavorable

tous les projets décidés « au-dessus » d'une collectivité ne peuvent lui être imputés. Ce principe me paraît tout à fait pertinent. En revanche, il me semble normal que l'artificialisation effectivement réalisée sur le périmètre des communes d'un SCoT soit, elle, mesurée et comptabilisée

se concentrant sur les zones souvent délaissées que sont les entrées de ville. Dans cette perspective, il vise à ce que les documents d'urbanisme garantissent la préservation des sols et la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.

les dispositions relatives à l'artificialisation des sols, notamment le moratoire commercial défini à l'article 52, inciteront les collectivités à repenser l'aménagement des entrées de ville. Cette mesure viendra compléter les dispositifs déjà mis en place pour permettre l'insertion urbaine et paysagère des aménagements en entrée de ville. On pense évidemment aux autorisations d'exploitation commerciale, aux opérations de revitalisation des territoires et au programme Petites Villes de demain. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable des PLU ne peut pas établir de dispositions prescriptives qui s'imposeraient aux autorisations d'urbanisme, telles que les auteurs de l'amendement le proposent. Le Gouvernement est donc défavorable

Une telle mention permettrait d'encourager la mutualisation des objectifs de consommation de l'espace au sein d'un PLUi sans pénaliser les communes rurales dans la répartition de ces objectifs, et de tenir compte des besoins de ces communes. économiques ? La commission estime que cette proposition fait doublon avec le droit existant. En effet, les PLU, comme tous les documents d'urbanisme, sont soumis aux principes généraux du code de l'urbanisme. Le préfet contrôle leur respect au moment de leur élaboration et peut même demander à ce qu'ils soient modifiés, au besoin pour

À ce titre, la sous-utilisation des sols dans les zones urbaines et l'existence de dents creuses doivent être combattues en détail, et le potentiel constructible établi par les PLU doit être utilisé à plein. Cet amendement a pour

économiques ? Cet amendement vise à donner au règlement des PLU la possibilité de forcer tous les propriétaires, dès qu'ils souhaitent construire sur leur terrain, à exploiter la totalité des droits à construire. Cela signifie concrètement qu'ils seraient contraints de bâtir le moindre centimètre carré autorisé par les règles d'urbanisme ou d'exploiter au maximum la hauteur autorisée, par

Il nous semble que la densification doit se faire des méthodes douces et qualitatives et garantir l'acceptabilité et l'adhésion des habitants. En outre, cette mesure est contre-productive : si le maire est tenu de refuser tous les projets qui ne maximisent pas la construction, plus personne ne souhaitera proposer de projets, et les parcelles resteront des friches. Enfin, à l'heure où nous parlons de nature en ville, d'îlots de chaleur, de qualité du cadre de vie, de végétalisation, souhaitons-nous vraiment forcer les Français à bétonner au maximum, à dire au revoir aux jardins et aux patios ? La commission est défavorable

de la qualité urbaine. Cette mesure impliquerait de construire sur l'emprise au sol maximale de la zone, quelle que soit la taille du terrain. Elle serait donc inapplicable pour certaines tailles de parcelle. Par ailleurs, elle ne permettrait pas de préserver des espaces de pleine terre. La densification, qui doit résulter d'un équilibre entre l'ambition des documents d'urbanisme et un dialogue entre les maîtres d'ouvrage et l'autorité compétente,

Je pense notamment au troisième objectif, celui d'« améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif ». L'objectif de régulation de l'artificialisation des sols ne doit pas reléguer les territoires ruraux au second plan de notre politique d'urbanisation. L'interprétation actuelle des lois rend quasi impossible toute construction en milieu rural : nous l'avons tous constaté dans nos intercommunalités lors de l'élaboration de certains PLUi. À l'heure où nos concitoyens souhaitent légitimement s'installer à la campagne, les territoires ruraux ne sont malheureusement pas en mesure de les accueillir.

Nous avons réécrit le dispositif de l'article 49 pour que celui-ci fasse explicitement mention des ZRR et des communes en perte démographique. En outre, les autres objectifs auxquels cet amendement fait référence, c'est-à-dire l'habitat, l'accès aux services et l'activité économique, sont explicitement inscrits aux articles 48 et 49.

ou d'une activité existant avant la promulgation de la présente loi, l'objectif étant de ne pas empêcher l'extension de projets industriels en cours ou à venir, et de les sécuriser.

d'une installation ou d'une activité existant avant la promulgation de la présente loi, lorsque cette extension intervient au sein d'une réserve foncière constituée avant cette même promulgation. Quel est l'avis de la commission des affaires

des extensions en continuité des espaces urbanisés ne soit pas calé sur la loi Littoral pour l'ensemble des communes et des intercommunalités qui n'y seraient pas soumises. La jurisprudence en la matière est en effet très particulière et n'est pas transposable en dehors des zones littorales.

Or certaines installations de production d'énergies renouvelables n'ont qu'une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol. Je pense notamment aux panneaux photovoltaïques

qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. En revanche, les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car elles accélèrent la déforestation. Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de dix ans prévue par le 1° du III de l'article 49, est légitime au vu de l'importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. À l'issue de cette période de dix ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l'article 48 permettra de traiter le cas des installations d'énergies renouvelables. La parole

elles. Pour les dix premières années, un dispositif fondé sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été prévu. Nous l'avons privilégié en raison de sa bonne appropriation par les territoires. Seulement, les panneaux photovoltaïques qui sont soumis à permis de construire seront par défaut comptabilisés comme de la consommation d'espace alors même que, selon les modalités techniques de pose, ils peuvent ne pas dégrader durablement les conditions écologiques des sols. Les amendements, qui visent à ne pas comptabiliser comme de la consommation d'espaces naturels les installations photovoltaïques réversibles qui n'affecteraient pas durablement les fonctions écologiques du sol, apparaissent donc tout à fait pertinents.

monsieur le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ? La commission, sous la houlette de notre présidente, a longuement débattu de ces sujets. Nous avons souhaité nous assurer que les mesures proposées ne faisaient pas peser une charge trop lourde sur les collectivités, que les délais fixés n'étaient pas irréalistes et, enfin, que le mécanisme en cascade fonctionnait. La commission estime que, si l'on veut faire des efforts ambitieux en faveur de la réduction de l'artificialisation, il est nécessaire que les documents d'urbanisme intègrent progressivement, et de manière différenciée, ces nouveaux objectifs. Il nous semble que l'équilibre obtenu

La commission a modifié ce dispositif pour prévoir que le conseil délibère sur l'opportunité d'engager la procédure d'évolution de ces documents. Nous proposons de supprimer une telle dérogation, qui nous paraît par trop imprécise et qui pourrait créer de fait une insécurité juridique. Les

même si cet amendement reprend les dispositions résultant des travaux de la commission, qui ont porté à trois ans le délai octroyé aux documents de planification pour intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation,

Les organisations professionnelles au sein du collège des professionnels du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ont pour rôle de formuler un avis sur l'ensemble des projets. Associer leurs représentants à l'élaboration de documents de planification ne me paraît pas opportun, dans la mesure où les objectifs qui seront définis portent davantage sur la programmation et la mixité sociale dans l'habitat, destinés à répondre aux besoins de la population, que sur la qualité de la construction,

Elle permet également de réduire le nombre de documents opposables aux SCoT. Cette ratification a donc une portée purement technique : elle permettra en particulier que l'ensemble des dispositions prévues à l'article 49 s'appliquent aux textes en vigueur. Quel est l'avis de la commission des affaires

économiques ? La compensation collective agricole prévoit, je le rappelle, que les porteurs de projets qui consomment des terres à vocation agricole doivent compenser la destruction des activités agricoles par des aides financières ou concrètes à la filière agricole locale.

d'ampleur, la procédure de l'étude préalable agricole et l'autorisation d'urbanisme sont deux démarches tout à fait distinctes. L'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers porte non pas sur le bien-fondé du projet, mais sur le contenu et la qualité de l'étude préalable agricole au regard de l'existence d'éventuels effets négatifs. Selon moi, le fait de conditionner l'autorisation d'urbanisme à l'avis conforme de cette commission sur cette étude serait une mesure une mesure disproportionnée. Par ailleurs, sans avoir recours au mécanisme de compensation collective, des dispositifs existent pour protéger les fonctionnalités agricoles, tels que les

me paraît pertinent que les CDPENAF, instances de dialogue utiles et impartiales, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées, si elles le souhaitent, sur tous les plans locaux d'urbanisme.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités et leurs regroupements dans la définition et la mise en oeuvre de leurs projets, notamment en matière de transition écologique et de développement économique.

qui évaluera le nombre de projets territoriaux accompagnés par l'ANCT et qui prendra en compte les transitions écologiques et énergétiques. Les missions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, telles qu'elles sont définies par la loi,

et impose, dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone tendue, la fixation d'une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable. Nous proposons la suppression de cet article, sachant que celle-ci n'empêchera pas les collectivités qui le souhaitent, en fonction de leurs besoins, de définir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

Nous avons notamment prévu que ce coefficient ne s'applique pas aux opérations menées sur des bâtiments existants, afin de répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées, notamment par les organismes de logement social. Nous avons aussi prévu que les surfaces végétalisées puissent être mutualisées à l'échelon d'un projet. La commission est donc défavorable

M. Frédéric Marchand. L'article 49 E impose, dans le cadre du PLU, une part minimale de surface en pleine terre végétalisée dans les espaces les plus denses de France, à savoir les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique. Afin d'adapter les exigences à

Je partage le souhait de clarifier le régime juridique des démarches de végétalisation de l'espace public, qui sont mises en place par certaines communes. Ce cadre législatif, qui relève des règles d'utilisation du domaine public et, plus spécifiquement, du régime des autorisations d'occupation temporaire,

débatte tous les trois ans, au lieu de tous les six ans, de l'adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d'urbanisme et d'aménagement. Prévoir un échange sur ce sujet majeur à mi-mandat plutôt qu'une fois tous les six ans nous paraît plus pertinent. Quel économiques ? Je rappelle tout d'abord que cette évaluation a été créée sur l'initiative de notre commission. Aujourd'hui, l'ensemble des documents d'urbanisme sont soumis à une évaluation périodique, à l'exception de la carte communale. Il nous a donc semblé pertinent de les inscrire aussi dans cette logique de bilan.

bilan, telle qu'elle existe aujourd'hui pour les PLU et les SCoT. Lors de l'examen en commission, nous avons introduit cet article pour organiser tous les six ans, au sein du conseil municipal, un débat portant sur l'adéquation entre les orientations de la politique d'urbanisme de la commune et sa carte communale. Nous constatons tous que certaines cartes communales datent parfois de plus de vingt Nul ne se pose plus la question de savoir si ces documents sont cohérents avec les enjeux actuels de la vie communale. Je rappelle qu'une telle évaluation existe déjà pour les PLU et les SCoT selon un format plus poussé et plus détaillé. Pour faire suite aux échanges que nous avons eus en commission, je vous propose ici de faire un pas supplémentaire dans cette en prévoyant que, comme pour les PLU et les SCoT, le conseil municipal délibère sur l'opportunité ou non de réviser la carte. Cette révision n'est bien sûr qu'une faculté, la commune restant souveraine. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le fait

À ce stade, la commission estime qu'il n'est pas opportun de modifier l'étendue de l'inventaire prévu. Les observatoires de l'habitat et du foncier sont surtout situés en zone tendue où la question la plus pressante est celle de la pénurie de logements. Bien sûr, il n'est pas inutile d'avoir des données plus importantes, mais nous ne souhaitons pas rendre l'inventaire des locaux économiques obligatoire. Alors que les observatoires existants se mettent tout juste en place, avec des moyens limités, et que le présent article prévoit déjà d'en étendre la portée, il me paraît prématuré d'élargir leurs missions à l'implantation d'activités

à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d'artificialisation des sols envisageable dans le cadre du projet global de territoire. Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d'une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation

dans la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est d'autant plus fondamental que ces derniers disposent des leviers pour la limiter : la délivrance des permis de construire, les décisions d'ouverture à l'urbanisation, la planification locale ou les politiques de préservation de certains espaces. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable

vise à exclure les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte de l'obligation d'établissement d'un rapport annuel sur l'artificialisation des sols. En effet, les territoires ultramarins

permettront une meilleure connaissance de ces phénomènes d'artificialisation. Ils peuvent donner l'occasion de faire valoir les spécificités ultramarines. De plus, comme nous l'avons souligné, ils ne feront pas peser une charge administrative trop importante sur les collectivités. La commission est donc défavorable

La commission ne souhaite pas transformer cette faculté en obligation. Elle privilégie une boîte à outils plutôt qu'une approche coercitive, et une densification douce et qualitative plutôt que quantitative. C'est d'ailleurs la philosophie de l'amendement de la commission, qui tend à créer une telle faculté

En l'état actuel du droit, il est déjà possible de fixer une densité minimale pour les projets qui se développent autour des transports en commun. Par ailleurs, toujours en vertu du droit en vigueur, le cahier des charges de cession des lots d'une ZAC, qui vise à définir la constructibilité autorisée, encadre d'ores et déjà étroitement les projets en prévoyant des prescriptions techniques urbaines et architecturales. Il peut donc porter sur la densité des constructions, dans le respect des règles qui sont fixées par les documents d'urbanisme.

économiques ? Je suis entièrement d'accord avec le principe avancé par M. Marchand : toute dérogation aux règles du PLU doit être expressément autorisée par le maire ou le président de l'EPCI compétent pour délivrer les permis, et le nombre de dérogations doit rester limité. C'est pourquoi, en commission, nous avons réécrit cet article pour supprimer le passage à un système de dérogations de droit, auxquelles le maire ne pourrait que difficilement s'opposer. L'article tel qu'il est rédigé aujourd'hui exige désormais l'accord de la commune ou de l'EPCI. En revanche, il me semble que la possibilité de recourir aux dérogations limitées dans les GOU et les ORT, et pas uniquement dans les zones denses, est une bonne chose.

L'article 51 A, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, visait à encourager la densification en zone tendue, en permettant que des dérogations

et la construction d'étages supplémentaires pour les bâtiments existants. Dans le système actuel, le maire doit motiver sa décision lorsqu'il accorde une dérogation pour transformer des bureaux.

un système de droit, sauf opposition. Toute dérogation au PLU doit être expressément autorisée par le maire ou le président d'EPCI compétent pour délivrer les permis, et le nombre de dérogations doit rester limité. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle souhaite

543 rectifié vise à préciser que les opérations de création ou d'agrandissement de logements, qui peuvent bénéficier de dérogations, incluent celles qui modifient les parties communes de ces logements ou leurs équipements, comme les cuisines communes, les buanderies ou les ventilations.

tend à opérer plusieurs modifications. Entre autres, il a pour objet de supprimer la possibilité, pour les projets de transformation de bâtiments en logements, de déroger exceptionnellement aux règles de mixité sociale. Je rappelle que nous avions collectivement voté cette dérogation en 2018, lors de l'examen de la loi portant La transformation d'un bâtiment préexistant implique de travailler avec un volume d'espace, un gabarit et des conditions prédéterminés. Elle peut donc concerner de petits bâtiments. L'application des quotas de logements sociaux sur de si petites opérations ne se justifie pas et serait contre-productive pour les opérations de transformation. En outre, cette dérogation est octroyée par la commune ou l'EPCI si jamais l'élu estime que les quotas de logements sociaux doivent s'appliquer et sont pertinents, il peut très facilement refuser une telle dérogation. Je rappelle aussi que cette dérogation aux règles de mixité sociale ne peut pas être délivrée dans les communes carencées en logement social. La commission En revanche, la commission est tout à fait favorable à l'amendement de repli n° 545 rectifié, qui tend à corriger une erreur de rédaction.

environnementale pour 2020 (RE2020) en matière de performance environnementale des constructions impliqueront un recours plus important aux constructions en bois. Or, dans certains cas, les règles de hauteur des PLU ne permettent pas d'autoriser des charpentes en bois dont le gabarit est plus important que les bâtiments environnants. Si l'on veut commencer dès aujourd'hui la transition du secteur du bâtiment et encourager l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, il est pertinent de prévoir une dérogation limitée aux règles des PLU. La commission émet donc

Concrètement, les planchers d'un immeuble ayant une structure en bois doivent avoir une épaisseur plus importante que des planchers en béton pour atteindre les mêmes performances acoustiques et énergétiques. Ces exigences seront encore plus contraignantes dans le cadre de la RE2020. Dans certains cas, la hauteur maximale définie par le PLU pourrait contraindre les constructions en bois à avoir un nombre d'étages inférieur à celui de constructions dotées d'une structure plus classique. Cela peut effectivement nuire à la viabilité économique des projets, mais aussi aller à l'encontre de l'objectif de densité fixé par le PLU.

Cet amendement a pour objet de soumettre certains projets, au moyen d'une procédure adaptée et en raison de leur dimensionnement, à une déclaration préalable en lieu et place d'un permis de construire.

Je suis favorable à un élargissement du champ de la déclaration préalable pour réduire les délais sur les projets les plus simples, mais à condition d'en garantir la qualité. Enfin, ces dispositions ont vocation à s'appliquer de façon uniforme sur tout le territoire, sous peine de créer une incertitude

à la rénovation et à la réhabilitation, à renvoyer de nombreux paramètres à un décret en Conseil d'État et à supprimer les dispositions visant à garantir que cette expérimentation soit instaurée sur l'initiative des communes qui le souhaitent.

En effet, depuis la loi ÉLAN, les EPCI à fiscalité propre peuvent adhérer à un EPF, tandis que les communes ne peuvent plus y adhérer de façon isolée. Dès lors, pour cet article, comme dans le passé lors de l'examen de la loi ÉLAN, la question se pose de rétablir l'équité. Dans un premier temps, il est nécessaire que l'EPCI délibère sur l'adhésion à l'EPFL puis, dans un second temps, en cas de refus de l'EPCI, que la commune puisse adhérer de manière individuelle.

économiques ? Effectivement, cette disposition figurait initialement dans le projet de loi 4D. Mais il serait regrettable de ne pas avancer au plus vite sur un sujet qui tient à coeur à de nombreuses communes qui, sans être la ville principale d'un EPCI, souhaiteraient néanmoins bénéficier d'une ORT, même si la ville principale ne subit pas de dévitalisation. Je le rappelle, une ORT permet de lutter, entre autres, contre la vacance commerciale et de réhabiliter des bâtiments. C'est un outil utile pour lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Il est donc judicieux de ne pas attendre inutilement pour renforcer les pouvoirs des communes en la matière. Le Gouvernement est défavorable

économiques ? Je ne pense pas qu'il soit opportun de supprimer cette étude, car elle permettra d'étudier la façon dont une opération d'aménagement peut être encore plus efficace que les règles de densité prévues par le SCoT. C'est donc au contraire un apport bienvenu. Je rappelle par ailleurs qu'elle ne s'applique qu'aux opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale, c'est-à-dire à celles qui sont réalisées par des porteurs de projets importants. Le Gouvernement est donc défavorable

le cadre de la construction des surfaces commerciales. En revanche, votre texte, madame la ministre, ne comporte aucune mesure comparable pour mieux réguler l'implantation des entrepôts de e-commerce. Si aucune évolution n'intervenait, comment pourrait-on l'expliquer

Nous sommes face à un modèle de développement qui influence directement l'aménagement de nos territoires, l'équité entre les acteurs économiques, notre modèle social et nos modes de consommation. Le gigantisme des infrastructures logistiques et la pression exercée sur les territoires doivent nous interpeller, d'autant que nous ne partons pas de rien : de nombreux travaux et études ont déjà été réalisés sur le sujet. Le récent rapport de nos collègues Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau esquisse des perspectives pour un développement plus durable des entrepôts de e-commerce. Avec mon groupe, nous proposons de confier de nouveaux outils Il s'agit, tout d'abord, de soumettre les entrepôts de e-commerce au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il faudrait aussi fixer une trajectoire pour conditionner, à court terme, les autorisations de construire à la desserte de ces entrepôts par des modes de transport massifiés et durables. Nous souhaitons que le texte adopté par le Sénat comprenne des avancées, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises.

des finances (IGF), un rééquilibrage fiscal et réglementaire rapide. Le développement fulgurant des géants du e-commerce va à l'encontre de l'objectif de relocalisation de notre économie. Il est tout d'abord destructeur pour l'emploi. Les conclusions de France Stratégie et de l'IGF sont sans appel : plus le commerce en ligne est fort dans un secteur, plus la baisse de l'emploi est marquée. Il est destructeur pour les droits des salariés, ainsi que pour le tissu économique et social du commerce de proximité et de la ruralité. Il est également destructeur pour les finances publiques, Amazon étant le roi de l'optimisation fiscale en Europe. Ce groupe ne paie ainsi aucun impôt sur les sociétés, pour un chiffre d'affaires pourtant estimé à 6,5 milliards d'euros

Elle n'est aujourd'hui pas satisfaisante, même s'il faut rappeler que le commerce représente moins de 5 % de l'artificialisation des sols. Pour autant, le n'est pas une option, car si l'impact en matière d'artificialisation des sols n'est pas majeur, il n'est pas inexistant non plus. C'est cette problématique qu'entend traiter l'article 52, qui prévoit l'interdiction de construire des surfaces commerciales de plus de 10 000 mètres carrés d'emprise au sol. Il s'agit d'un renforcement inédit, unique de la réglementation commerciale. En commission, nous sommes parvenus à un équilibre qui permet à la fois de limiter l'implantation de ces grandes surfaces, de redonner le pouvoir de décision aux acteurs locaux et de favoriser la respiration du parc commercial. Nous nous sommes ainsi assurés que les extensions de bâtiments ne soient pas interdites, sous réserve que leur emprise au sol soit faible extension soit permise par bâtiment. Nous avons également remplacé la notion de surface de vente par celle d'emprise au sol, puisque la surface de vente ne dit absolument rien de l'artificialisation des sols qu'un projet peut engendrer.

mystérieusement absent du projet de loi, je pense, comme presque tout le monde, qu'il est temps de nous pencher enfin sur l'implantation parfois désordonnée de ces infrastructures trop longtemps absentes des radars de la réglementation. Leur impact sur l'environnement et sur les équilibres territoriaux, qu'il soit positif ou négatif, est réel, et il faut en tenir compte. Je proposerai donc un amendement qui vise à soumettre la création des entrepôts de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher à autorisation.

au modèle des grandes zones commerciales, qui défigurent nos entrées de ville et contribuent à dévitaliser nos coeurs de ville et nos commerces de proximité. Nous faisons un pas décisif pour limiter l'étalement urbain, préserver la vitalité de nos sols et réduire notre consommation d'espace. À compter de la promulgation de la loi, il sera interdit de construire, en artificialisant les sols, de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 mètres carrés. Nous limitons donc le développement de ce qu'on appelle des « boîtes à chaussures » en périphérie des communes et de nos lieux de vie. C'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat : de la Convention citoyenne pour le climat : comme elle, nous pensons nécessaire de prévoir des cas où il est possible de déroger à cette interdiction générale pour l'adapter à la diversité des territoires. Nous avons exclu qu'une dérogation puisse être accordée pour un projet d'une surface de vente de 10 000 mètres

En ce qui concerne les entrepôts logistiques, il me semble qu'il faut séparer deux grandes questions de nature sensiblement différente : d'un côté, la place du e-commerce dans nos modes de consommation, la concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne, et la place des grands acteurs du numérique dans le e-commerce ; de l'autre, l'aménagement de l'espace dans la lutte contre l'artificialisation des sols et le rôle des entrepôts et des très grands entrepôts en la matière. Les entrepôts de e-commerce ne représentent actuellement que moins de 1 % des surfaces artificialisées sur le territoire. Ils ne constituent donc pas, dans les faits, un énorme gisement de consommation d'espace à résorber. Bien sûr, ces entrepôts peuvent avoir localement un impact significatif mais, dans les faits, il est parfois difficile de savoir si un entrepôt est utilisé ou pas par les plateformes de commerce en ligne. Certains servent à la fois à l'entreposage du commerce physique et à la vente en ligne. nationale a adopté un amendement du rapporteur, qui vise à renforcer le contrôle de l'implantation des activités logistiques dans les documents d'urbanisme. Plusieurs amendements ont pour objet de mieux prendre en compte l'artificialisation des sols et la consommation d'espace par les entrepôts. Tout cela me semble apporter une réponse proportionnée proportionnée aux enjeux, en complément des mesures générales et ambitieuses que nous prenons pour lutter contre l'artificialisation des sols. Nous pourrons ainsi davantage orienter l'implantation des entrepôts sur des friches et limiter leur emprise au sol.

Nous proposons d'avancer dans trois directions. La première, c'est de soumettre à autorisation d'exploitation commerciale la création, l'extension ou la transformation d'un bâtiment en entrepôt logistique d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement

est établie au regard des besoins du territoire, de l'absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches, et de la continuité du projet avec le type d'urbanisation du secteur et le tissu urbain existant,

un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l'extension ou la transformation d'un bâtiment existant en entrepôt logistique d'une surface supérieure à 3 000 mètres carrés. La parole est

telles que Amazon ou encore Alibaba, est dévastateur. C'est la raison pour laquelle des mesures fortes doivent être prises. L'article issu des travaux de la commission ne nous satisfait pas, car il ne permet pas, à ce stade, de réguler la croissance exceptionnelle des géants du e-commerce.

camions par jour. Devons-nous continuer à accepter cette « amazonisation » de la France, cette destruction inévitable du tissu du commerce de proximité et de tous les liens sociaux qui font la vie quotidienne des bourgs et des centres-villes ? stopper cette logique mortifère de concurrence déloyale pour prendre, enfin, des décisions d'intérêt général, bonnes pour l'emploi et l'activité économique des TPE et PME, pour l'aménagement du territoire et pour l'environnement ? Madame la ministre, j'ai bien entendu que les multinationales du e-commerce cherchaient à brouiller les cartes en utilisant des entrepôts qui ne sont pas complètement dédiés au stockage ou au e-commerce, mais il ne faut pas les laisser faire ! Je pense que nous pouvons trouver un large consensus sur cette question au sein

Il me semble qu'une telle mesure est exagérément restrictive et qu'elle conduirait à figer le secteur du commerce en l'état, ce qui aurait de nombreux effets de bord. Premièrement, elle conduirait à octroyer une rente ... Exact ! ... à tous les commerces déjà installés, qui n'auraient alors plus aucune concurrence à craindre. Deuxièmement, cela reviendrait à ignorer que tous les acteurs commerciaux ne sont pas encore véritablement parvenus à maturité.

force est de reconnaître que la technique impose ses règles et que le consommateur accédera nécessairement, plus ou moins rapidement, et quelle que soit la législation, à toutes les formes de distribution.

souligné le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis du 27 janvier dernier relatif à ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à une autorisation d'exploitation commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d'application de l'article

la surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a permis de ne pas être soumis aux règles d'implantation du code de commerce. Or il représente aujourd'hui plus de 20 % dans certains secteurs, tels l'électronique, le textile ou les produits culturels.

Il s'agit en outre de prendre en compte la surface de vente et celle du parc de stationnement affecté au local commercial, lequel artificialise aussi grandement les sols. Par ailleurs, la notion d'emprise au sol, adoptée en commission, ne peut être suffisante pour lutter contre l'ensemble des externalités néfastes des implantations des zones commerciales.

Cette dernière est en effet sans lien direct avec l'artificialisation des sols, dès lors que les surfaces de vente peuvent s'empiler au sein d'un même bâtiment à étages. Cette disposition permettra d'intégrer les ensembles commerciaux non concernés par la définition précédente, malgré la volonté affichée du rapporteur pour avis, afin d'autoriser la densification des centres commerciaux, sans limite de surface, en incitant à diminuer l'emprise au sol des parcs de stationnement.

à quelques projets particulièrement visibles et en permettant bien trop de dérogations. Ainsi, le gros de l'artificialisation provoquée par les surfaces commerciales de périphérie affecté, dans un moment où les locaux commerciaux souffrent d'un taux de vacance très important, encore aggravé par la crise économique et sanitaire, et où le développement des commerces de centre-ville et des petits commerces souffre profondément. Il faut

j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur, une délégation du Sénat de la République de Pologne et du Bundesrat de la République fédérale d'Allemagne. l'invitation des groupes d'amitié France-Allemagne et France-Pologne, nos collègues allemands et polonais ont participé, cet après-midi, à la conférence consacrée au trentième anniversaire du « triangle de Weimar », placée sous le haut patronage du président du Sénat. Les travaux portaient principalement sur les perspectives d'avenir de la diplomatie européenne dans le cadre du triangle germano-franco-polonais de Weimar, ainsi que sur les nouveaux défis à relever ensemble en matière de défense. La délégation polonaise, en visite en France pour quelques jours, est conduite par le président du groupe Pologne-France, Aleksander Pociej. Elle est accompagnée par notre collègue Valérie Boyer, présidente du groupe d'amitié France-Pologne. La délégation allemande est conduite par M. Tobias Hans, président du groupe d'amitié franco-allemande du Bundesrat, ministre-président de Sarre. Elle est accompagnée par notre collègue Ronan Le Gleut, président du groupe d'amitié France-Allemagne. Nous souhaitons à nos collègues allemands et polonais la plus cordiale bienvenue au Sénat français

M. Daniel Salmon. En l'état, les dispositions des alinéas 7 à 12 de l'article 52 autorisent de nombreuses dérogations, qui vident de leur substance les dispositions de cet article et en affaiblissent la portée.

Les habitants des territoires concernés n'attendent pas forcément de nouveaux centres commerciaux de près de 10 000 mètres carrés. Quant aux dérogations pouvant être accordées aux « opérations d'aménagement » visant à « favoriser [ ...] la mixité fonctionnelle », c'est la porte ouverte à l'autorisation de presque tous les projets.

de friches commerciales, artisanales ou industrielles est possible dans l'enveloppe urbaine existante. Il est en effet urgent, d'une part, d'empêcher le recours à de nouvelles terres agricoles et, d'autre part, de créer des dispositifs favorisant la réutilisation et la restructuration des friches dans la perspective de nouvelles dynamiques commerciales.

Cette disposition précise que les autorisations d'exploitation commerciale ayant un impact sur l'artificialisation des sols ne peuvent être délivrées à titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des solutions de substitution et mené une réflexion détaillée

Il est nécessaire de fixer les conditions de la compensation pour la rendre effective. Cette proposition permet de mettre en place un mécanisme spécifique inspiré de la compensation en matière de défrichement, tout en assurant de bénéficier des avantages du cadrage établi

y compris ceux qui constituent une richesse pour notre patrimoine, comme c'est le cas des zones AOC. Il est possible de concevoir un certain nombre d'aménagements avec le texte tel qu'il est rédigé.

Cet amendement vise à apporter une clarification sur les dérogations au principe de l'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales.

le CESE estime que la séquence ERC est quelque peu bafouée dans la mesure où l'on s'attache à compenser sans avoir préalablement cherché à éviter et à réduire. Cet amendement vise ainsi à préciser que les autorisations d'exploitation commerciale ayant un impact sur l'artificialisation des sols ne peuvent être délivrées, à titre dérogatoire, que si le pétitionnaire a recherché des options de remplacement et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l'impact, mais d'abord, et prioritairement, sur les mesures permettant d'éviter et de réduire l'impact de l'artificialisation. Il tend également à fixer les conditions de la compensation

Elle permet de limiter la surcapacité e-commerciale afin de protéger les emplois des commerces physiques déjà menacés ainsi que l'empreinte carbone liée à nos importations et de préserver les sols naturels et agricoles. Le seuil de 3 000 mètres carrés nous paraît constituer un bon compromis : il permet d'ouvrir la voie au développement de petits entrepôts de e-commerce à destination des commerces locaux ou d'activités de vente en ligne d'articles de seconde main en France. l'objectif n'est pas de nuire au commerce en ligne, mais de réguler enfin les géants du secteur, toujours exemptés des contraintes que l'on impose à tous les autres. Oui, il convient de mettre un coup d'arrêt à ces implantations anarchiques, de favoriser leur sobriété environnementale et d'optimiser l'utilisation d'infrastructures existantes : proximité des gares, livraison au dernier kilomètre, reconversion de friches industrielles. Il convient aussi de donner aux commerces de proximité le temps de développer des offres commerciales collectives, physiques ou utilisant les services numériques adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs. Les

Certaines d'entre elles s'engagent dans une course aux délais de livraison pour des biens qui, dans la plupart des cas, sont produits à des milliers de kilomètres. Le commerce de détail des biens vendus à distance a ainsi connu une hausse de 37 % en 2020 par rapport à 2019. Or la surcapacité des commerces en ligne contribue à la dévitalisation des bourgs-centres et accroît l'empreinte carbone de la France liée aux importations de produits et à l'augmentation du flux de marchandises. comporte des risques pour les emplois des commerces physiques, mais aussi pour l'emploi tout court, en raison de l'automatisation du travail dans ses entrepôts. En outre, l'installation d'entrepôts logistiques participe à l'étalement urbain et constitue une menace pour les sols naturels et agricoles.

ce qui permettra d'organiser une concertation entre élus, commerçants, grandes entreprises de e-commerce et aménageurs pour parvenir à un modèle sain pour l'environnement et pour l'emploi.

pour des surfaces de vente et non pour des surfaces de e-commerce. Le Gouvernement continue de travailler sur la place du e-commerce tant du point de vue environnemental que dans l'équilibre global du commerce, y compris sur les sujets d'égalité et d'équité dans la taxation. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

prévoit que le préfet pourra désormais se référer aux enjeux de gestion économe des sols pour accorder ou non une autorisation ICPE, il nous semble que cette disposition n'est pas assez ambitieuse : d'une part, le préfet ne sera pas tenu d'en tenir compte ; d'autre part, le régime applicable aux entrepôts a été assoupli depuis la loi du Cette évolution est une bonne chose pour l'attractivité de notre territoire, mais il nous semble que de fortes interrogations persistent dans le cas spécifique des entrepôts du commerce en ligne. Au demeurant, l'absence de réglementation commerciale entourant l'installation de ces entrepôts peut s'apparenter à une distorsion de concurrence vis-à-vis des commerçants physiques, dont l'implantation est soumise à un corpus étoffé de règles. Or si les entrepôts logistiques traditionnels sont généralement de simples maillons dans la chaîne d'approvisionnement, ce ne semble pas être le cas des entrepôts de commerce en ligne, qui se rapprochent davantage de la notion de centres de distribution en bout de chaîne. Cet amendement vise à proposer que les entrepôts principalement dédiés au commerce en ligne soient soumis à autorisation d'exploitation commerciale lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres

Si la réutilisation de ces lieux participe à la poursuite de l'objectif « zéro artificialisation nette », le conditionnement de l'autorisation commerciale au type de sol sur lequel s'implante l'entrepôt de e-commerce est une erreur à double titre. ce n'est pas juridiquement pertinent, l'autorisation commerciale devant être délivrée en fonction de la nature de l'activité et non du sol sur lequel elle s'implante

Redon-Sarrazy. Les auteurs de cet amendement proposent de corriger l'inégalité de traitement entre commerce physique et e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Une telle mesure avait été adoptée au Sénat lors des débats sur la loi du

il faut favoriser une planification stratégique des plateformes logistiques au niveau local. Il s'agir de faciliter la localisation d'entrepôts et de plateformes multimodales dans des lieux pertinents, si possible à proximité d'axes de transport massifiés tels que les points d'arrivée de trains ou de barges. Alors que les entrepôts se sont déployés par le passé autour de corridors logistiques, leur implantation tend, depuis dix ans, à se développer à proximité des grandes villes, en particulier les grandes métropoles françaises. Sous l'effet de la montée en puissance du e-commerce, on observe une hausse de la surface moyenne des bâtiments et une localisation de plus en plus proche des bassins de consommation. Dans l'objectif de lutter contre l'artificialisation, il faut mettre en place des critères de sélectivité : les bons projets sont ceux qui sont desservis par un ou deux modes de transport autres que la route. Notre amendement vise à conditionner toute nouvelle implantation d'entrepôt ou extension à des conditions de desserte par des modes massifiés et durables de transports définis par décret en conseil d'État. Ce décret devra prendre en compte l'objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises

pour s'assurer que les obligations, notamment en vue d'atteindre l'objectif du « zéro artificialisation », sont respectées.

Monsieur Genet, l'artificialisation pour la construction de parcs de stationnement dans les dix prochaines années, par rapport aux dix années écoulées. Or l'État n'est pas le seul constructeur de ces parcs de stationnement. Par ailleurs, l'installation

doit également concerner les nouveaux parkings et ne peut se réduire uniquement à l'existant. La végétalisation de l'ensemble des parkings et des aires de stationnement est un objectif majeur pour favoriser la biodiversité et lutter contre les effets du changement climatique.

les ombrières sur les parkings. Nous nous réjouissons de l'adoption de l'amendement n° 2092 à l'article 24, qui favorise l'implantation de procédés d'énergies renouvelables sur les ombrières des parkings,

qui traite de l'intégration des enjeux logistiques au sein du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique. Quel

Les nouvelles exigences normatives fixées par cet article sont disproportionnées par rapport aux objectifs du projet de loi. Nous proposons d'alléger ces exigences en laissant aux intercommunalités à fiscalité propre, gestionnaires des zones d'activité, le soin de déterminer la manière de procéder à leur inventaire et d'évaluer les enjeux de requalification ou de mutation des zones. Cet amendement tend ainsi à rendre plus réaliste et plus soutenable l'obligation nouvelle imposée aux collectivités. Les deux

pour servir la cause de l'arrêt de l'artificialisation des terres et définir les opportunités existantes afin de favoriser la réalisation d'installations ferroviaires de desserte terminale.

vise donc à développer le flux de marchandises vers ces espaces nouveaux.

Cet amendement tend à proposer que l'inventaire prévu par l'article 53 identifie les opportunités de créer les installations terminales embranchées à même de favoriser une desserte non routière de ces zones d'activité.

Cette servitude ouvre aux propriétaires un droit de délaissement leur permettant d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé de procéder à son acquisition.

la dynamique « zéro artificialisation nette » va très certainement renchérir le prix du foncier, renforcer les logiques de relégation du logement social là où les terrains sont moins chers et réduire les capacités de construire du logement social. Cela affectera nécessairement la répartition géographique et renforcera les inégalités territoriales. Toutes les opportunités de recyclage du foncier doivent être mobilisées au service du logement social.

l'amendement n° 964 rectifié La commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, dont cet amendement est issu, ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d'aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches.

a dressé le constat du manque d'informations sur l'état des territoires, notamment en ce qui concerne les friches. Elle a préconisé l'adoption d'une véritable politique nationale en la matière, ainsi qu'une grande loi sur les sols. En effet, vouloir aménager durablement un sol pollué est un non-sens total. C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête a orienté ses travaux en vue de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d'aménagement durable. Mais le défaut d'inventaire exhaustif nous empêche

sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) la création et l'animation d'un réseau national des inventaires de friches, d'octroi d'aides financières à destination des gérants d'inventaire de friches, ainsi qu'un rôle de conseil auprès de l'État, des collectivités ou des autres gérants d'inventaire. La parole est

dans le cas où le maire souhaite augmenter le nombre de lots par rapport au nombre prévu initialement, afin d'autoriser les subdivisions. Cela permet ainsi un meilleur équilibre entre un objectif de densification, qui est celui de la collectivité, et le maintien des droits et obligations des membres du lotissement

est à M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à identifier les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l'urbanisation. À l'heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées. Il apparaît ainsi difficile de savoir quelle surface elles occupent faute de base de données suffisante et fiable. Cet amendement vise donc à pallier un tel manque de connaissances en inscrivant le recensement des friches dans les missions affectées aux établissements publics fonciers. Nous proposons également que ces friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du plan local d'urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d'aménagement. Quel

de l'amendement est déjà satisfaite par l'article 49 du projet de loi, qui confie aux établissements publics fonciers la mission d'assister les observatoires de l'habitat et du foncier dans le recensement des friches et impose au règlement du PLU d'identifier et de délimiter les friches. La nouvelle obligation envisagée disproportionnée au vu des travaux de recensement déjà prévus par le texte en matière de friches. Par ailleurs, cela ne me semble pas être le bon vecteur. Le règlement de PLU sert à décliner des normes d'urbanisme par secteur, et non à réaliser des inventaires. Cela obligerait chaque commune et EPCI à réviser son

Le développement de la cyclo-mobilité professionnelle des entreprises, dont celles de cyclo-logistique, suppose d'offrir du foncier accessible et bien situé pour être à portée d'intervention de la clientèle et pour assurer de bonnes conditions de repos aux personnels. personnels. Selon leur situation dans le tissu urbain, les friches représentent souvent une bonne opportunité d'affecter et d'aménager de l'espace urbain à destination d'entreprises ayant fait le choix d'une mobilité durable. La logistique urbaine du dernier kilomètre constitue un défi considérable pour les territoires urbains et les acteurs de la logistique. Génératrice d'embouteillages, avec 20 % du trafic automobile, d'émission de gaz à effet de serre- 15 % des émissions de CO2 sont dues au transport de marchandises -, de pollution de l'air, soit 30 % de la pollution en ville, et de nuisances sonores, la logistique est pourtant indispensable au bon fonctionnement des villes. La cyclo-logistique est une réponse durable à l'essor de la livraison et aux émissions de gaz à effet de serre qui l'accompagnent. Propre, silencieuse et limitant l'encombrement, elle se substitue avec efficacité aux véhicules utilitaires légers.

ou de distribution des friches. Sur le fond, l'amendement vise à donner priorité aux « projets inscrits dans une démarche durable » sans toutefois les définir ou donner le moindre critère. Seul l'usage du vélo est mentionné. Il ne me paraît pas souhaitable d'accorder ainsi une priorité particulière au vélo, qui ne se prête pas à tous les types d'activités.

des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d'« usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l'« usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec

Nous proposons ainsi de définir précisément la notion et les différentes catégories d'usage retenues en matière de sites et sols pollués. La définition serait plus proche de celle d'un bien commun que de celle d'un bien économique.

des sols ». Son article 3 définit la notion d'usage en matière de sites et sols pollués. En effet, actuellement, le principe de gestion du risque par l'usage qui sous-tend l'approche française en matière de sites et sols pollués ne peut s'appuyer sur aucune définition claire des notions d'usage, de remise en état ou de réhabilitation. Les travaux de notre commission d'enquête, tous courants politiques confondus, démontré la nécessité de clarifier ces notions-clés sous peine de laisser une marge d'interprétation trop importante à la jurisprudence et aux maîtres d'ouvrage. Il est donc temps de mettre un terme à une telle insécurité juridique. De surcroît, la notion d'usage est fondamentale, car elle définit le niveau de risque à prendre en compte et ainsi le niveau de pollution acceptable et les mesures de dépollution nécessaires. Cependant, elle ne fait pas l'objet d'une définition spécifique. Fixer une telle typologie permettrait en outre de faciliter le travail de contrôle et de prescription de l'administration

d'enquête : « Nous devons donc rentrer dans ces débats au niveau des clauses et des contrats, ce qui génère beaucoup de contentieux : quel site, à quel endroit, quel type de pollution, quel sera l'usage ... Nous nous dirigeons aujourd'hui vers un " droit mou " jurisprudentiel, sauf si un texte intervient pour mettre en place un " droit dur "

me paraît déjà satisfaite par un projet de décret d'application de l'article 57 de la loi ASAP, qui prévoit de définir l'usage et la réhabilitation au niveau réglementaire. Le projet de décret, en cours d'examen par le Conseil d'État, devrait être publié dans les prochaines semaines. Je demande donc le retrait de ces amendements

des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en secteur d'information sur les sols (SIS) ou sur les terrains d'anciennes ICPE.

de prévoir l'obligation pour le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage d'un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt et réhabilitée de transmettre au préfet un mémoire de réhabilitation. Le représentant de l'État se prononce sur ce mémoire, qui détaille les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état projeté des sols. Il est en effet anormal que l'administration ne puisse contrôler de manière effective les attestations d'études des sols établies par les bureaux d'études.

comme pour l'eau et l'air. La question de la surveillance des mesures de gestion pour les sites situés en secteur d'information des sols ou sur les terrains d'anciennes ICPE Les inspecteurs des installations classées ont un rôle absolument mineur dans le contrôle et la surveillance de la qualité des travaux effectués sur ces sites. C'est, ma foi, fort étonnant. Le code de l'environnement prévoit prévoit une obligation de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution, mais en renvoyant le contrôle de cette obligation à des bureaux d'études certifiés par le biais d'une attestation. C'est très léger. D'abord, cela ne permet pas à l'administration de contrôler l'effectivité des mesures de gestion, ni leur pertinence. Là aussi, c'est étonnant. Ensuite, des pièces fournies par des bureaux d'études ne permettent pas de détecter des insuffisances dans la réhabilitation. Cet amendement vise à renforcer le rôle de l'administration, en l'occurrence la Dreal, et à instaurer une base de données permettant une meilleure information en matière de réhabilitation des sols, ainsi que des mesures de remédiation compatible du sol avec son usage futur envisagé. La Dreal serait ainsi chargée d'analyser les données des bureaux d'études et de délivrer l'attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de gestion. La parole

encadrant la remise en état et la réhabilitation des sites. Seule la méthodologie de 2017, qui est dépourvue de réelle valeur juridique, décrit aujourd'hui les bonnes pratiques compilées par l'administration. Nous ne sommes pas en train de dire que les bureaux d'études sont laxistes. Mais le déficit de contrôle et d'encadrement peut conduire à opter pour des solutions peu souhaitables sur le plan environnemental. Nous voulons donc doter l'administration d'une compétence de contrôle de la mise en oeuvre des obligations de diagnostic ou des mesures de gestion de la pollution, même quand elles sont attestées par un bureau d'études, en cas de doute sur leur qualité ou leur réalisation concrète. À

suite des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l'article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d'évolution ». L'attestation de réalisation de l'étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d'ouvrage, qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information. L'intérêt et la finalité d'une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, mais serait seulement transmis pour information au préfet de département, restent flous et contestables. Au-delà, une telle étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu'aucun intérêt opérationnel ne soit démontré. L'article 54 s'inscrit donc en totale contradiction avec l'objectif de simplification administrative et d'allégement des procédures visé par le Gouvernement. Il est ainsi proposé de le supprimer. Bacchi, pour présenter l'amendement n° 203. L'article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d'ouvrage un outil d'aide à la décision lors de la conception d'un projet de construction, de démolition ou d'aménagement leur permettant d'identifier les potentiels de réversibilité et d'évolution des bâtiments concernés par l'opération. Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, les maîtres d'ouvrage devront alors réaliser une étude de potentiel de réversibilité du bâtiment adossée au diagnostic déchets dans le cas de démolition. Cette action est déjà réalisée par les maîtres d'ouvrage professionnels. De plus, cette nouvelle disposition occasionne de nouvelles dépenses, largement sans objet, coûteuses et sans possibilité d'amortissement. En effet, l'étude risque d'être insuffisante pour constituer une véritable aide à la décision. En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d'effet réel sur la consommation de ressources naturelles. L'article 54 a reçu un accueil unanimement défavorable de la part du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. La parole

de quelle manière le bâtiment pourrait être transformé et remodelé pour accueillir de nouveaux types d'activités au cours de sa vie. À titre personnel, je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette étude, car le cycle de vie d'un bâtiment est si long que l'état des techniques au moment de sa construction ne permet pas d'imaginer son potentiel d'évolution cinquante ans plus tard. les démolitions concernent, dans la majeure partie des cas, des bâtiments très dégradés ou ne correspondant plus aux attentes. Je crains donc que cette nouvelle étude préalable ne termine, comme d'autres, dans des tiroirs dont elle ne sortira jamais et ne trouve pas d'application concrète. Quel usage en fera l'administration ? De surcroît, son coût ne sera pas négligeable pour les constructeurs. Pour autant, la question de la transformation des bâtiments est importante au regard de la quantité de gaz à effet de serre et de déchets générés par le secteur de la construction. Il faut effectivement encourager le réemploi des bâtiments et leur conception durable. En commission, nous avions décidé de ne pas amender cet article, afin de pouvoir en débattre collectivement en séance publique. Pour cette raison, et au regard des différents arguments pour et contre, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.

qui impose de réaliser une étude sur les possibilités d'évolution des bâtiments, traduit la volonté de la Convention citoyenne pour le climat de privilégier les rénovations plutôt que les démolitions suivies de reconstruction. L'approche choisie par le Gouvernement, fidèle à la demande des citoyens, est incitative. Elle vise à sensibiliser les maîtres d'ouvrage à l'importance de concevoir des constructions neuves, qui anticipent et facilitent les rénovations futures. Certains d'entre eux le font déjà, et il convient de généraliser cette bonne pratique. Un décret viendra préciser les constructions visées par cet article. Ce seront nécessairement les projets les plus importants,

cette disposition, qui permet de lutter contre les dépôts sauvages de déchets du bâtiment et d'assurer une meilleure traçabilité des matériaux. Un problème d'articulation de l'entrée en vigueur d'une ordonnance a eu pour effet de supprimer la disposition du code correspondant. Le présent article vise uniquement à la réintégrer audit code. En conséquence, l'avis est défavorable.

Les grandes filières économiques, les grands groupes sociaux et culturels n'ont pas encore appréhendé la rapidité et l'importance du dérèglement climatique.

La séance est reprise. Nous allons donc procéder à la seconde délibération de l'article 68. Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement

la version issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il s'agit de remplacer l'alinéa relatif à la pollution des sols par un alinéa qui fait référence au non-respect de la réglementation applicable aux déchets. En effet, la protection des sols sols n'est plus limitée au seul cas de pollution causée par des déchets ; elle recouvre un champ beaucoup plus vaste de pratiques agricoles qu'il convient de sécuriser juridiquement. Même amendé

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

heures trente. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription du projet de loi de finances rectificative pour 2021 à l'ordre du jour du mercredi 30 juin 2021, le soir, à la suite du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets se tiendront mardi